La numérisation des formalités pour la création, la modification et la cessation des entreprises implique que les futurs chefs d'entreprise soient mieux formés aux outils informatiques, ce qu'exigent également leurs relations numériques avec les clients et les différentes administrations. Il est donc nécessaire de mettre en place un stage spécifique de formation à l'outil informatique et digital. Quel

à Mme Nathalie Delattre. Les alinéas 3 et 4 du présent article ont été ajoutés en commission spéciale. Ils conduisent à complexifier de façon excessive les modalités de déroulement du stage, en distinguant une première et une seconde partie, dont le contenu, ambitieux, nécessiterait plus que la durée prévue, qui est de quelques jours. Il semble au contraire nécessaire de s'en tenir,, à une formation fondamentale, notamment en comptabilité, les autres types de formation éventuels n'ayant pas besoin d'être détaillés au niveau de la loi. Par ailleurs, le dispositif mis en place n'est pas contraignant alors qu'il s'adresse à des publics n'ayant aucune formation, puisque ceux qui ont bénéficié d'une formation au moins équivalente ou d'une expérience professionnelle sont dispensés de suivre le stage d'accompagnement à l'installation. C'est pourquoi il est proposé de supprimer ces alinéas.

avant son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises. La commission a précisé le contenu de la formation à effectuer sur une journée dans le mois qui suit l'immatriculation. Cependant, au regard de la densité de ce contenu, nous proposons que le stage soit de quatre jours, cette durée étant fractionnable, pour la première partie, qui est la plus précise et la plus fournie,

et à la comptabilité analytique, l'autre partie pouvant éventuellement être fractionnée. S'il paraît cohérent que la seconde partie du stage puisse intervenir dans les six mois suivant l'immatriculation, il paraît indispensable, en revanche, que la première partie de la formation intervienne obligatoirement avant l'immatriculation,

puisqu'il favorise la pérennité de certaines entreprises, l'argument du coût a également été beaucoup utilisé. Ainsi, modifier voire supprimer le stage de préparation à l'installation constituerait « une source d'allégements financiers pour les entrepreneurs concernés,

Pourtant, dans le même temps, le plafonnement du prix de ce stage, prévu par le droit en vigueur, est remis en cause par le texte de la commission.

dont nous ne connaissons pas la nature, « l'accompagnement de ceux qui s'installent et qui auraient besoin de compétences en matière de gestion » serait développé, mais à des prix non encadrés. Il y a là, selon nous, une certaine contradiction, pour ne pas dire incohérence. Et il semble bien que cet article n'a pour pour objet que de libéraliser l'offre de formation et d'assurer la croissance des sociétés de formation, et non celle des artisans. Aussi, pour éviter une libéralisation complète des offres de formation,

Cet amendement vise à revenir sur la position de la commission, qui a souhaité que le prix maximal du stage soit désormais fixé par l'APCMA,

: La parole est à M. Maurice Antiste. Les stages de formation sont indispensables aux entrepreneurs, en particulier à ceux qui s'installent. Ces stages doivent donc être renforcés, rendus gratuits, et certains modules doivent impérativement être traités.

connaissance des différents types de crédits qui leur seront proposés et des conditions d'accès à ces crédits, afin d'être en mesure de planifier au mieux le développement de leur activité.

De fait, la suppression de cette taxe implique la suppression de ce fonds, dont l'objet était de contribuer au financement d'actions de promotion et de communication à caractère national en faveur de l'artisanat. Or ce dispositif de mutualisation est pleinement voulu par les artisans, car il s'agit du seul moyen pour leur entreprise d'accéder à une communication grand public d'envergure : depuis sa création en 1997, ce fonds a contribué à installer durablement, dans l'esprit du public, une image positive de l'artisanat et une valorisation essentielle de ses métiers. Il a permis de stimuler l'orientation des jeunes vers l'apprentissage et l'emploi dans l'artisanat. C'est aussi grâce à ce dispositif que l'artisanat est aujourd'hui reconnu par une majorité des Français comme « la première entreprise de France L'article 5 vise à garantir la pérennité du principe de mutualisation, auquel les représentants de l'artisanat sont attachés. Le mécanisme de substitution proposé est compatible avec les règles du droit européen et reposera sur une contribution privée, portée par un organisme privé. Le présent amendement a pour objet de spécifier que les organisations visées doivent faire la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l'artisanat, et que l'accord est réputé valide y compris y compris dans le cas où une seule organisation professionnelle d'employeurs intéressée par l'artisanat et reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en serait signataire. La parole

Cette taxe provient d'une majoration de 10 % de la taxe pour frais de chambres de métiers et représente une contribution de 11 euros par an pour chaque entreprise artisanale. La suppression de cette taxe emporte la suppression du FNPCA, dont l'objet est de contribuer au financement d'actions de promotion et de communication à caractère national en faveur de l'artisanat. ce dispositif de mutualisation est pleinement voulu par les artisans, car il s'agit du seul moyen pour leur entreprise d'accéder à une communication grand public d'envergure depuis sa création en 1997, le FNPCA a contribué à installer durablement, dans l'esprit du public, une image positive de l'artisanat et une valorisation essentielle de ses métiers. Il a permis de stimuler l'orientation des jeunes vers l'apprentissage et l'emploi dans l'artisanat. C'est d'ailleurs grâce à ce dispositif que l'artisanat est aujourd'hui reconnu par une majorité des Français comme « la première entreprise de France Le présent amendement a pour objet d'accompagner ces évolutions en spécifiant que les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel doivent faire la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l'artisanat, et que l'accord est réputé valide y compris dans le cas où une seule organisation professionnelle d'employeurs intéressée par l'artisanat et reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en serait signataire. Quel est l'avis de la commission ? Il est difficile d'accepter qu'une seule organisation professionnelle d'employeurs, fût-elle très représentative de la profession d'artisan, puisse à elle seule mettre en place un régime de contribution volontaire obligatoire pour l'ensemble des entreprises artisanales. Aussi, l'avis est défavorable sur ces amendements. Monsieur le ministre,

l'amendement n° 188. L'article 5 du projet de loi introduit diverses dispositions en vue de clarifier et de simplifier le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée,

essentielles de l'EIRL. D'une part, la protection du patrimoine privé de l'entreprise au-delà de la seule insaisissabilité de la résidence principale, déjà accordée, permet d'affecter à l'activité professionnelle de l'entrepreneur un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. Cela le met à l'abri de certaines pressions bancaires au moment de faire l'inventaire de l'entreprise. D'autre part, nous voulons ouvrir la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés sans pour autant subir la charge administrative du formalisme lié à la forme sociétaire.

de droit de leur résidence principale sans aucune démarche à effectuer. On pourrait également imaginer en complément une évolution du régime fiscal de l'entrepreneur individuel, pour le rendre plus avantageux, sans recourir à l'EIRL.

d'autre part, la sanction de faillite personnelle lorsque l'EIRL a disposé des biens de son patrimoine professionnel comme s'ils étaient compris dans son patrimoine personnel sans intention frauduleuse. Il s'agit donc de simplifier la

774. Outre la correction de deux erreurs matérielles et deux coordinations, l'amendement n° 930 vise à mieux articuler la disposition selon laquelle le dépôt du bilan de l'EIRL auprès du registre de publicité légale dont il relève vaut actualisation de la composition de son patrimoine affecté et la possibilité, instaurée par le projet

auteurs de l'amendement n° 774 proposent de revenir sur plusieurs modifications qui ont été adoptées par la commission

? Je suis très favorable à l'amendement présenté par Julien Bargeton, qui vise à renforcer les droits du conjoint collaborateur, notamment sur les indemnités journalières. Le sujet est très concret.

l'avis de la commission

deux points auxquels les sénateurs devraient être sensibles. Nous avons étendu le statut de conjoint collaborateur salarié par défaut aux commerçants, aux artisans et aux professions libérales. C'est un élément de protection majeure du conjoint collaborateur, qui est souvent une femme.

Au nom de l'affection profonde que je porte au monde agricole- vous connaissez mon attachement aux paysans français ! -et au nom de la justice, il vous est proposé d'étendre ce statut de conjoint collaborateur salarié par défaut au monde agricole.

90 % des cas de femmes, pourra être couverte par une protection sociale adaptée, un régime de retraite et tous les avantages allant avec le statut de conjoint collaborateur salarié par défaut

il sera simple d'établir la preuve d'une activité constante auprès du conjoint dans une activité agricole et compliqué

amènera les entreprises à ne plus avoir d'obligation d'élaborer un règlement intérieur avec les salariés. Or le règlement intérieur est indispensable dans la relation entre le chef d'entreprise, les actionnaires- c'est rare, mais cela peut arriver

Quand on dénombre 199 seuils répartis sur 49 niveaux pour les PME, avec des méthodes de calcul multiples suivant qu'il s'agisse du code du travail, du code de commerce ou du code de la sécurité sociale,

le nombre de seuils fixés à 20 salariés est réduit, plusieurs seuils sont relevés de 20 à 50 salariés pour le taux réduit de la contribution au Fonds national d'aide au logement, ou FNAL, pour l'exonération de participation à l'effort de construction et pour l'absence d'obligation d'un règlement intérieur dans l'établissement, tandis que d'autres sont relevés de 200 à 250 salariés. nous avons entendu les remarques des acteurs économiques qui nous entourent. Il est enfin temps de leur offrir les souplesses nécessaires pour libérer les initiatives et les possibilités de développement et de supprimer un certain nombre de freins-

un effectif non stabilisé. J'espère que nos échanges dans cette assemblée auront pour unique objectif d'acter cette indispensable simplification, qui n'a que trop tardé. La parole est à M. Fabien Gay,

Pour vous donner un ordre de grandeur, un demi-millième de PIB représente la somme de 1,25 milliard d'euros, soit la production nationale de notre pays pendant un peu plus de 4 heures.

l'embauche ! L'argument, déjà avancé en 2014 par François Rebsamen, lequel avait prôné un gel des seuils sociaux pendant trois ans, revient aujourd'hui en force, tout comme celui, intimement lié, du coût excessif de la représentation du personnel en France. Dans son rapport de mars 2011 sur les relations industrielles en Europe, la Commission européenne avait effectué une étude comparative des attributions des instances représentatives du personnel au sein des différents États membres, en fonction des pouvoirs qui leur sont attribués. Sur la base d'une notation de 1 à 10, la France, avec 7 points, figurait dans le quatrième groupe de pays, derrière les pays scandinaves- Danemark en tête -, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche. Dans une note de 2011, l'INSEE, montrait que les effets sur l'emploi seraient marginaux : « En l'absence de seuils dans la législation, la proportion d'entreprises entre 0 et 9 salariés diminuerait de 0,4 point, tandis qu'elle augmenterait de 0,2 point dans chacune des tranches de 10 à 19 salariés et de 20 à 249 salariés

terrible ! Dans le monde contemporain, ce dont nous avons besoin, c'est qu'un dialogue social s'opère avec les salariés, que leurs droits soient reconnus et que l'on puisse réfléchir collectivement à l'avenir de l'entreprise, avec une juste répartition des richesses, des emplois et des investissements.

certaines obligations ne s'appliquant qu'aux entreprises ayant dépassé un certain seuil d'effectif. Il retient donc les seuils de 11, 50 et 250 salariés. De plus, il faudrait désormais que les seuils d'effectif soient franchis pendant cinq années consécutives pour que les obligations liées à ces seuils s'appliquent. La suppression du seuil de 20 salariés aura des conséquences concrètes sur la politique du logement social. La participation à l'effort de construction Action logement et le Fonds national d'aide au logement sera, par la suppression de ce seuil, uniquement due par les entreprises de plus de 50 salariés,

qui simplifie les mesures disparates du droit en vigueur dans les différents codes- cette harmonisation concernerait un quart des 199 obligations recensées actuellement dans différentes réglementations ; l'instauration de la règle de franchissement du seuil des cinq ans, qui aura des conséquences positives à court terme en lissant les effets de seuil ; le relèvement de 20 à 50 salariés du seuil d'assujettissement à la participation employeur à l'effort de construction et au taux normal de la contribution au FNAL.

ainsi, redonner du souffle à notre économie ! Je pense strictement l'inverse ! Je pense qu'un pacte social, avec une juste représentation des salariés et leur association à un certain nombre de décisions d'avenir, est la seule façon de redresser l'économie nationale.

C'est bien la preuve que la politique économique que nous menons, avec le Président de la République, avec le Premier ministre, avec la majorité, donne des résultats. En la matière, seuls les chiffres comptent : au cours des trente : au cours des trente dernières années, les niveaux de chômage les plus bas ont été atteints vers les années 2000 et 2001, à la fin des années Jospin,

Et je suis convaincu que ces mesures relatives aux seuils permettront de créer de l'emploi pour les Français et pour leurs enfants. Elles seules ne suffiront pas, bien entendu, il n'y a pas de potion magique, et il faut développer la formation, les qualifications,

est intégralement compensée, je vous rassure, à la fois par une taxe affectée et par des dotations budgétaires. Quant au FNAL, et je reviens vers Jacques Mézard, nous avons fait le choix d'une taxe affectée pour créer ce dynamisme nécessaire dont Action Logement avait besoin.

dispose, d'une part, que les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale du travail- cela revient à avoir un raisonnement équivalent au temps plein -, d'autre part, que les salariés titulaires d'un CDD ou qui sont mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu., dans les autres cas, ces salariés sont comptabilisés. Ces dispositions ont vocation à demeurer et sont plus précises que ce qui est proposé

Il est en effet prévu que le passage au seuil supérieur ne soit pris en considération qu'à condition que l'augmentation des effectifs se maintienne pendant cinq années consécutives. Et chaque année où l'effectif repasserait en dessous du seuil entraînerait le redémarrage du décompte. Cette règle donne une marge de manoeuvre de manoeuvre assez importante aux entreprises et leur laisse la possibilité de développer des stratégies sur plusieurs années. En jouant avec les effectifs, elles pourraient parfaitement s'assurer de remettre le décompte à zéro, afin de ne jamais dépasser un seuil et, par conséquent, de ne pas avoir à respecter leurs obligations légales. une telle mesure laisse la porte ouverte à des abus, mais elle a des conséquences fiscales et sociales de plus en plus importantes. Ce délai de cinq ans repousse en effet l'assujettissement des entreprises à leur obligation fiscale, pour un coût estimé par l'étude d'impact à 500 millions d'euros par an. Encore une fois, le Gouvernement fait peser sur la sécurité sociale le coût des politiques en faveur de l'entreprise. Nous ne pouvons l'accepter ! C'est pourquoi nous présentons cet amendement, qui tend à modifier la règle de prise en compte du franchissement d'un seuil. Nous proposons que le passage au seuil supérieur soit pris en considération lorsque celui-ci est dépassé pendant douze mois, consécutifs ou non, sur une durée de trois ans. Cette période de douze mois permet de s'assurer que la hausse d'effectifs est pérenne, mais ces douze mois n'ont pas à être consécutifs et sont étalés sur trois ans, ce qui permet aussi d'empêcher les éventuelles stratégies d'évitement que pourraient mettre en place les entreprises. De plus, et enfin, le lissage sur trois ans limite l'incidence fiscale de cette mesure. L'amendement

avant les ordonnances Travail de 2017. Je suis d'autant plus défavorable à cet amendement que je pense que le risque d'abus de la part d'entreprises jouant sur leurs effectifs

est en train de tout défaire, on nous répond : « Circulez braves gens, parlementaires, sénatrices et sénateurs, il n'y a rien à craindre : tout est sous contrôle du Gouvernement

Mensonge ! Vous dites que nous attaquons le droit syndical, la représentation des salariés, ... Vous l'avez déjà fait ! ... vous pouvez monter sur vos grands chevaux, mais ce n'est pas la vérité. Or je veux rétablir la vérité. Je revendique la politique économique que nous menons, mais je ne veux pas qu'on nous fasse porter le chapeau d'une politique économique qui ne serait pas la nôtre.

non pas sur les peurs que peuvent susciter certains propos.

Alors, de deux choses l'une : soit vous n'avez pas lu le texte, soit vous voulez induire les Français en erreur. Dans les deux cas, ce n'est pas recommandable ! S'agissant des représentants du personnel,

si vous me cherchez sur mon texte que défend l'actuelle majorité, vous me trouverez. Mais je ne laisserai jamais affirmer des contre-vérités sur un texte soumis au vote du législateur, parce que ce n'est pas ma conception de la démocratie. J'admets parfaitement que, dans nos discussions, M. Gay et moi-même ayons des conceptions radicalement différentes de l'économie, de l'entreprise, des PME, des chefs d'entreprise, de la place des salariés, des syndicats, des instances représentatives du personnel. Mais que vous décriviez mal le texte qui est soumis à votre examen et à votre vote, je ne laisserai pas passer cela ! S'il faut des dizaines d'heures de discussions et de négociations entre nous jusqu'à faire émerger la vérité, nous en passerons par là. J'ai tout mon temps et j'ai toute la patience nécessaire.

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions remettant en cause le compromis pris en compte dans la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, à savoir que les entreprises de moins 50 salariés peuvent être qualifiées d'artisanales et que, au-delà, le droit de suite ne s'applique plus. Cet amendement a également pour objet d'éviter la multiplication du nombre d'entreprises doubles ressortissantes des chambres de commerce et d'industrie, d'une part, et des chambres de métiers et de l'artisanat, d'autre part, sous peine de conduire inévitablement à la fusion des deux réseaux consulaires. Il tend aussi à éviter la création de services d'accompagnement des entreprises qui seraient redondants dans les réseaux consulaires, dans un contexte de restrictions budgétaires et de recherche de plus de mutualisations des actions prévues par le projet de loi, notamment aux articles 13 B et 13 C. Enfin, cet amendement vise à assurer une cohérence entre les différents articles du projet de loi PACTE. L'article 2 prévoyant la création d'un registre général des entreprises, avec une fusion à terme du registre du commerce et des sociétés avec le répertoire des métiers notamment, il n'est pas opportun de complexifier les dispositifs liés à ces registres pour un temps qui sera nécessairement limité. La parole est à Mme Nathalie Delattre,

de mettre à disposition, dans une entreprise, un local syndical. Cette mesure a été supprimée par l'Assemblée nationale, puis rétablie par notre commission spéciale. Si les entreprises estiment que le dialogue social

par les services de santé au travail. Le suivi de l'état de santé des travailleurs doit se faire autour d'une personne physique, quels que soient la nature du contrat et le nombre d'heures de travail. On ne saurait imaginer une prise en charge médicale partielle sous prétexte qu'une personne ne travaille pas à temps plein. ne travaille pas à temps plein. Or la Cour de cassation vient d'introduire, hors contexte, un critère relatif au temps de travail dans la définition de l'effectif à prendre en compte par les services de santé au travail, notamment pour le calcul des cotisations. décision renforce l'ambiguïté déjà introduite par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, appliqués au suivi de la santé. De plus, si l'effectif de l'entreprise est calculé sur la base de ces deux articles, les apprentis et certains salariés employés à durée déterminée sont exclus du calcul de l'effectif.

à élargir les modalités actuelles de décompte des salariés qui se fondent notamment sur la nature du contrat et sur la durée du travail du salarié, en particulier pour la détermination de la cotisation de l'entreprise ont donc deux conséquences : elles écrasent l'harmonisation en matière d'appréciation des seuils, prévue à l'alinéa 57 pour la seule obligation de mise à jour du document d'adhésion au service de santé au travail, et elles augmentent fortement les cotisations employeur au SSTI.

Le Président de la République a annoncé son intention de faire du handicap l'une des priorités du quinquennat, et la question de l'emploi des personnes en situation du handicap est bel et bien essentielle. Le présent projet de loi maintient le seuil d'effectif à 20 salariés pour le déclenchement de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés,

Mais je considère que la logique d'harmonisation et de lissage du droit en matière d'appréciation et de franchissement des seuils est bonne : elle doit s'appliquer à cette obligation. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié la règle de calcul de l'OETH,

? Cet amendement tend à appliquer, à l'aide versée par l'État à l'employeur dans les entreprises de moins de 250 salariés qui ont signé des contrats d'apprentissage, les nouvelles règles d'appréciation et et de franchissement des seuils d'effectifs. L'aide à l'apprentissage ne serait donc plus versée dès que l'entreprise franchit le seuil de 250 salariés, en moyenne, pendant un an. La commission spéciale

le ministre. Cet amendement a pour objet les dispositions transitoires nécessaires pour que les anciens dispositifs de gel ou de lissage du taux de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continuent à s'appliquer à leurs bénéficiaires actuels.

les obligations associées sont également des formes de la socialisation des besoins et des ressources qui a fait notre système social. Par exemple, les entreprises qui augmentent leur effectif au-delà de 20 salariés doivent s'acquitter d'une participation à l'effort de construction

C'est le 1 % qui a permis la réalisation de la plupart des quatre millions de logements sociaux dans notre pays, réponse aux besoins collectifs particulièrement prégnants en ce domaine.

on peut effectivement assécher la ressource et décider, en toute conscience, de laisser les mal-logés et les sans-abri aux prises avec l'état actuel du marché, lequel est dérégulé depuis plus de trente

toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, pendant toute la durée de son application. Or, à compter de 2019, l'État ne compensera pas la baisse du forfait social. C'est, hélas !, ce qui a été voté

mise au point. Je mets aux voix l'article 6, modifié. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est presque minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à minuit et demi, afin d'aller plus avant dans l'examen de ce texte.

C'est plutôt ironique, quand on sait que le Gouvernement affiche comme objectif l'harmonisation de l'ensemble des seuils ... À travers cet article, la modification des seuils est encore l'occasion de porter atteinte aux droits des salariés. En effet, il est prévu de relever à 100 tous les seuils fixés à 50 salariés dans le code du travail. Autrement dit, toutes les entreprises comprenant entre 50 et 99 salariés seraient soudainement exonérées d'une multitude d'obligations. En droit du travail, le seuil de 50 salariés est central. Il entraîne l'application de règles dans des dans des domaines variés. Il en est ainsi du droit du travail collectif, qui encadre la représentation des salariés dans l'entreprise. Ce droit à représentation serait mis à mal, puisque la réunion d'un comité social et économique disposant de l'intégralité de ses attributions serait reportée, tout comme l'obligation de nommer des délégués syndicaux centraux d'entreprise et d'établissement. Ces derniers verraient d'ailleurs leurs heures de délégation réduites, alors même que ce temps est nécessaire à l'exercice de leurs attributions. ont une autre conséquence notable, quant au licenciement pour motif économique. Les entreprises doivent démontrer des difficultés économiques, dont la durée dépend de la taille de l'entreprise. La démonstration du licenciement serait facilitée, puisque les entreprises comptant entre 50 et 99 salariés n'auraient à faire état que de deux trimestres de difficultés, contre trois actuellement. on pourrait également citer la durée du travail, la formation professionnelle, la santé, la sécurité et les conditions de travail. Une fois de plus, nous nous opposons à ce que les mesures de simplification soient l'occasion de porter atteinte aux droits des salariés. Nous sommes tout à fait favorables à une harmonisation des droits des salariés, à condition qu'elle soit créatrice de droits. Comme ce n'est pas le cas de cet article, nous vous présentons cet amendement de suppression. La parole

le projet de loi PACTE prévoyant déjà, en son article 6, un délai de cinq ans pendant lesquels les obligations liées au passage d'un seuil à un autre ne s'appliquent pas.

La dernière réforme du code du travail, issue des ordonnances de septembre 2017, a renforcé ce seuil en y attachant près d'une quinzaine d'obligations déclenchées auparavant à 20 salariés.

Le coût d'un emploi supplémentaire ne se résume pas au coût marginal du dernier salarié arrivé. D'un point de vue psychologique, enfin, le changement de dimension lié à l'adaptation de la structure de l'entreprise peut faire craindre au dirigeant une perte de contrôle. Les économistes

le code du travail. Que chacun mesure bien ce qu'il va voter et le message qu'il va adresser à tous les salariés français et à toutes les organisations syndicales : cette disposition concerne le licenciement économique,

Le scrutin est ouvert.

Cet amendement vise à rétablir la gouvernance de Business France telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale. Quel est l'avis de la commission

Dans un contexte difficile pour nombre de nos concitoyens, du fait de salaires peu élevés ou gelés et, en même temps, d'une hausse des prix, le moment des soldes peut être crucial, car il permet de se vêtir, voire de vêtir sa famille, sans se ruiner. Pour autant, les soldes ne peuvent être considérés comme une aide aux ménages modestes : ils ne doivent pas devenir l'arbre qui cache la forêt, nous empêchant de voir que le véritable problème

Nous en arrivons même à inventer des vêtements jetables, bons à n'être portés qu'une fois ! Alors que partout les ressources s'amenuisent, l'utilisation de coton gourmand en eau, des polyesters et autres dérivés du pétrole, les vêtements assemblés dans plusieurs pays et les stocks acheminés à travers la planète et détruits lorsqu'ils ne sont pas vendus doivent nous conduire à nous interroger : quel modèle de société voulons-nous encourager Une société du toujours plus vite jetable, donc du déchet à outrance, avec une infime partie seulement des déchets recyclés à grands coûts énergétiques, ou une société plus durable, plus responsable et respectueuse de la planète

La parole est à M. Pierre Louault. Cet amendement vise à fixer une durée maximale et non une période déterminée de soldes, afin de préserver la liberté des commerçants. Si les soldes demeurent un événement très attendu, le sentiment d'urgence qu'ils ont pu susciter par le passé a disparu, les pratiques ayant évolué. Il est donc souhaitable de réduire leur durée maximale.

favorables ! Dans les régions et départements d'outre-mer, la saisonnalité des ventes et les périodes touristiques ne sont évidemment pas les mêmes que dans l'Hexagone.

Compte tenu des délais d'adoption du projet de loi, la mesure ne prendrait effet, au mieux, qu'aux soldes d'hiver de janvier 2020. Son application immédiate, proposée par les auteurs de l'amendement, rendrait possible la mise en place du nouveau régime dès les soldes d'été de 2019. Il faut néanmoins être attentif au petit commerce et lui laisser un temps suffisant pour adapter ses stocks. Si nous adoptons la loi en mars ou en avril, je ne suis pas certaine que le délai sera suffisant pour les soldes de juillet prochain.

Le délai retenu pour l'entrée en vigueur de la mesure sur les soldes doit permettre aux commerçants de s'adapter, notamment pour leurs approvisionnements et leurs ventes. Issu de la concertation sur les soldes tenue à l'automne dernier, il tient compte des contraintes de la négociation et des spécificités de gestion de stocks des commerces indépendants. La réforme des soldes envisagée s'inscrit dans une démarche de revitalisation commerciale des centres-villes, en particulier dans les villes moyennes.